La séance est reprise.

Madame la présidente, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, nous examinons cet après midi le projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024.

la nature même de notre tissu économique, mais également, en cette année particulière, à l’effet des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qu’il ne faut pas sous estimer.

Dans son avis, le Haut Conseil des finances publiques estime que les prévisions de croissance et d’inflation retenues dans le PLFG sont « réalistes » et que notre prévision de déficit est « plausible

d’environ 50 milliards d’euros est principalement lié à l’évolution des prélèvements obligatoires, dont le produit est revu à la baisse pour plus de 40 milliards d’euros par rapport aux prévisions initiales ; ce chiffre s’explique pour moitié par l’exécution constatée en 2023.

vous. L’écart par rapport à la prévision initiale résulte également du dynamisme des dépenses publiques en 2024, en dépit, je tiens à le rappeler, des efforts de freinage bien réels enclenchés par le précédent gouvernement en matière de dépense de l’État – j’y reviendrai.

Nous avons travaillé en particulier avec la commission des affaires sociales dans le cadre de l’examen du PLFSS, afin de réagir le plus rapidement possible. Nous proposons de mobiliser plusieurs leviers qui permettront de ramener à 0,2 milliard d’euros le dépassement par rapport à la trajectoire de l’Ondam 2025 présentée dans le texte

Qu’il s’agisse de l’État, de la sécurité sociale ou des collectivités, nous sommes tous soumis aux difficultés de prévision et de gestion qu’impliquent les périodes de crise puis de rebond économique, comme celles que nous avons connues au cours des deux derniers exercices. notre niveau d’endettement actuel résulte moins de ces aléas que des choix collectifs que nous avons faits ces dernières années. Je le répète régulièrement, si nous avons protégé notre pays lors des crises, il est aujourd’hui de notre responsabilité collective de redresser nos comptes, dans un contexte où l’endettement a évidemment largement augmenté.

Ces annulations portent très majoritairement sur la réserve de précaution, renforcée cet été grâce au surgel de juillet que je viens d’évoquer. Elles ont fait l’objet de discussions approfondies avec l’ensemble des ministères, tout comme les ouvertures de crédits que je vous présenterai dans instant. Ce travail utile et nécessaire de construction collective nous a permis de calibrer les moyens au plus près des besoins réels de gestion des administrations, en limitant les crédits au strict nécessaire.

mais aussi à la prise en charge des forces de l’ordre et de défense mobilisées pour assurer la sécurité sur place, ou encore aux mesures de soutien aux entreprises, aux salariés, aux collectivités et aux hôpitaux, qui permettent à la Nouvelle Calédonie de tenir. Au total, 1 milliard d’euros de dépenses supplémentaires sont prévus en 2024 à ce titre.

Il s’agit également de compléter le financement des dépenses de guichet en faveur des plus vulnérables, dépenses dont le niveau, vous le savez, peut varier en cours de gestion. Concrètement, il est ici question des bourses sur critères sociaux pour les étudiants, de l’allocation aux adultes handicapés, de la préservation du parc d’hébergement d’urgence ou encore de l’accueil des réfugiés ukrainiens.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, c’est la seconde fois que nous examinons un projet de loi de finances de fin de gestion. En effet,

Les raisons du rejet ne me sont pas apparues clairement, autant le dire. De nouveau, le Sénat va donc avoir à se prononcer sur la copie initiale du Gouvernement et il nous reviendra, en commission mixte paritaire, de tout faire pour nous mettre d’accord avec les députés sur un texte

dans la moyenne des prévisions du Consensus des économistes et parfaitement en ligne avec les prévisions « institutionnelles ». Cette prévision est d’autant plus crédible à mes yeux que, selon les dernières données de l’Insee, l’acquis de croissance au troisième trimestre est déjà de 1,1 %.

souligne, les facteurs de croissance n’ont rien à voir avec ce qui était anticipé, en tout cas par le précédent gouvernement. La croissance devait être tirée par la consommation. Or elle a été soutenue non seulement par le commerce extérieur, mais aussi et surtout par la demande publique. En clair, c’est le dérapage complet du déficit public cette année qui a permis d’atteindre l’objectif de croissance du Gouvernement, fixé à 1,1 %. J’entends nombre de responsables politiques se féliciter de ladite croissance. Pourtant, je n’avais pas cru entendre ni comprendre que l’explosion du déficit était au cœur de la politique économique portée par le ou les précédents gouvernements. Le fait est donc là malgré l’atteinte de la prévision de croissance pour 2024, la situation des finances publiques s’est encore très fortement dégradée pour dépasser le niveau historique de 2023.

Comme je l’ai indiqué ici même ce matin, je regrette toujours et à ce stade que personne n’assume la responsabilité politique de ce dérapage et de cette sortie de route. J’en viens au présent projet de loi de fin de gestion. Nous l’avons également indiqué dans le cadre de notre mission sur la dégradation des finances publiques, la principale cause de la dégradation se situe du côté des recettes. recettes. La prévision de croissance retenue dans le PLF pour 2024 était tout bonnement surévaluée : 1,4 % au lieu de 1,1 % de croissance réalisée. S’y ajoute une prévision d’élasticité des prélèvements obligatoires à la croissance que l’on peut qualifier de très, voire trop, optimiste

net de crédits de paiement. L’an dernier, j’avais, ici, qualifié le projet de loi de fin de gestion de texte « riche, voire opulent ». Cette année, on en revient, et c’est salutaire, à davantage de mesure.

ni exagéré ni, pour répondre à mes collègues de gauche, la marque d’une austérité brutale : c’est une réponse, partielle, à la dégradation – à l’aggravation – de la situation des finances publiques, donc à la chute des recettes. tel résultat est relativement facile à atteindre, nous l’avions souligné dans nos travaux sur le projet de loi de finances pour 2024 : à l’époque, souvenez vous, toutes les missions du budget de l’État étaient en progression, à part la mission « Anciens combattants, Le point de départ des crédits de la loi de finances pour 2024 était donc très haut. Il était même trop haut. Ce texte marque une autre rupture par rapport aux années précédentes : c’est la première fois depuis 2019 et la quatrième fois en treize ans que les annulations de crédits dépassent les ouvertures de crédits dans le collectif budgétaire de fin d’année. Les ouvertures de crédit les plus importantes concernent, pour les citer très rapidement, les dépenses supplémentaires

Sur la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances », ce sont les surcoûts des prestations sociales, en l’occurrence l’aide aux adultes handicapés (AAH) et l’aide universelle d’urgence pour les personnes victimes de violences conjugales, qui justifient à titre principal les ouvertures de crédits. Parmi les missions dont les crédits sont globalement en diminution, la mission « Investir pour la France de 2030 » fait l’objet d’une annulation très importante de crédits, de 1,2 milliard justifiée par le lissage de la trésorerie des opérateurs. Cela rejoint l’analyse faite par notre rapporteur spécial, Laurent Somon. Sur la mission « Engagements financiers de l’État », je relève que le reflux de l’inflation permet de réduire la charge de la dette de 537 millions d’euros par rapport à la prévision. Habituellement, le projet de loi de fin de gestion prévoit des augmentations d’emplois. Il n’y en a pas cette année : le plafond des autorisations d’emplois n’est pas majoré. Je veux y voir également le signe d’un retour à une gestion plus

troublée notamment par le refus du gouvernement précédent de présenter un projet de loi de finances rectificative. Nous le redisons, je le redis, seul un PLFR aurait permis, plus tôt et en temps utile, de redresser la barre

Je vous propose que nous restions sur la même ligne, de façon à veiller au respect de l’autorisation parlementaire accordée en loi de finances initiale. le texte ne contient aucune surprise, puisqu’il repose sur le même scénario que le projet de loi de finances pour 2025 : une croissance prévue à 1,1 % en 2024 et une inflation contenue à 2,1 %. Nous notons que ces prévisions ont été jugées réalistes par le Haut Conseil des finances publiques. Pour ce qui est du déficit, si nous voulons redresser nos finances publiques, il est impératif de le contenir à 6,1 % du PIB en 2024. Cette étape est indispensable pour atteindre les 5 % en 2025 et viser

de près de 6 milliards d’euros par rapport à la loi de finances initiale pour 2024. Ce redressement progressif est un préalable nécessaire si nous voulons garantir la soutenabilité de nos finances publiques ; il y va de notre responsabilité.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce budget supplémentaire est un objet législatif encore nouveau et peu connu des Français.

De 49.3 en 49.3, le Gouvernement avait alors fait le choix de contourner le débat parlementaire et d’ignorer les alertes citoyennes, sociales et syndicales quant à la situation du pays. Quelques mois plus tard, le 24 février 2024, il annonçait, sans aucun débat démocratique, une coupe de 10 milliards d’euros dans le financement des services publics. C’était bien la démonstration que ses prévisions étaient fausses et que le budget était insincère

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de loi de finances de fin de gestion est le deuxième du genre présenté au Parlement, à la suite de la modification en 2021 de la fameuse loi organique relative aux lois de finances. Cette évolution émane d’une initiative parlementaire dont vous êtes l’auteur, monsieur Saint Martin.

L’an dernier, les recettes fiscales de l’impôt sur le revenu ont été surestimées de près de 8 milliards d’euros à moins de deux mois de la fin de l’exercice. Les ministres de l’époque le savaient. Un projet de loi de finances rectificative aurait dû être l’occasion de redresser la barre et d’ajuster les recettes ; il n’en fut rien.

Nous savons maintenant que le PLF pour 2024 était insincère. Dès le mois de février dernier et la publication d’un décret d’annulation des crédits, la détérioration brutale du solde public nécessitait un projet de loi de finances rectificative. hormis les soutiens du Président de la République – et encore : Bruno Le Maire en réclamait un lui même ! –, chacun convenait qu’il n’y avait pas d’autre solution, y compris vos nouveaux alliés de la majorité sénatoriale. Votre rapport sur ce PLFG, monsieur le rapporteur général, ne dit pas autre chose. Si le déficit a

vision dogmatique de l’économie, dont la politique de l’offre constitue le seul horizon, en arrive à déstabiliser jusqu’à vos alliés du parti Les Républicains. Même pour eux, l’ampleur des dépenses fiscales non compensées semble excessive, d’autant que ce projet de loi de finances de fin de gestion confirme l’échec économique et, surtout, la catastrophe financière provoqués par cet entêtement : 6,1 % de déficit hors période de crise, 163 milliards d’euros, alors même que tous les leviers possibles de réduction des dépenses ont été actionnés – décret d’annulation de crédits, gel, surgel –, désormais confirmés par ce texte.

s’avère d’autant plus navrante que les ressources actuellement mobilisées pour le maintien de l’ordre auraient pu être mieux employées à réduire les inégalités persistantes entre les Kanaks, les Caldoches et les autres communautés. Quant au coût de la dissolution de l’Assemblée nationale, qui a dû être supporté sans compensation par les collectivités, le Président de la République en porte l’entière responsabilité. Au chapitre des collectivités, justement, le compte n’y est pas. Nous ne pouvons que déplorer l’absence dans ce texte de compensation des décisions de l’État relatives aux départements, notamment l’extension du Ségur

des débats ! Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires votera contre ce projet de loi de finances de fin de gestion, qui conforte la trajectoire prise par le Gouvernement avant les élections législatives

en tout cas inédit. Présenté comme un simple ajustement technique, le projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024 est en réalité révélateur des carences et des erreurs de la politique budgétaire des exécutifs ces dernières années. Depuis sept ans, les gouvernements successifs ont tous fait le choix de sacrifier les recettes fiscales sur l’autel de l’idéologie néolibérale, affaiblissant ainsi les capacités de l’État à faire face aux différentes crises. Les réductions d’impôts mises en œuvre depuis 2017 ont engendré un manque à gagner global d’environ 62 milliards d’euros par an. Cette diminution des ressources fiscales a eu plusieurs conséquences notables.

Ce débat dépasse les frontières de l’arithmétique budgétaire : il touche au cœur même de la justice sociale et de la soutenabilité économique de notre modèle. La situation que je viens d’exposer est la conséquence directe d’une politique marquée par des prévisions irréalistes et par des décisions irresponsables. Dès décembre 2023, le Gouvernement disposait de notes internes alarmantes sur la dégradation des finances publiques. Pourtant, aucune mesure corrective sérieuse n’a été prise.

« pari » politique risqué combiné à un « déni » des réalités économiques et budgétaires. Face à une situation budgétaire critique, le Gouvernement aurait dû présenter un projet de loi de finances rectificative dès le premier semestre 2024, comme le groupe socialiste le demandait. Un tel texte aurait permis d’engager les ajustements nécessaires pour contenir le déficit.

Ces ex ténors du Gouvernement ont qualifié le rapport de notre commission de « réquisitoire d’opposants politiques, truffé de mensonges ». Cette réaction est non seulement injustifiée, mais elle témoigne surtout de leur fébrilité et de leur volonté de discréditer une assemblée qui a le défaut de ne pas être d’accord avec eux. Le rapport sénatorial repose sur des données factuelles et sur des analyses précises, loin des déclarations péremptoires.

Pour reprendre l’expression de l’économiste Michaël Zemmour, la logique du Gouvernement est marquée par ce que l’on pourrait qualifier de « néolibéralisme de la stagnation La logique austéritaire qui sous tend ce PLFG est non seulement injuste, mais aussi contre productive. Investir dans la transition écologique, renforcer nos services publics, voilà ce qui stimulerait l’économie tout en préparant notre pays aux défis de demain À l’inverse, persister dans cette logique d’austérité ne fera qu’aggraver les fractures sociales et territoriales. Mes chers collègues, ce PLFG n’est pas un simple texte technique il symbolise une politique budgétaire et fiscale à la fois injuste et inefficace. Malgré le dépôt par le rapporteur général, dont je tiens à saluer la persévérance sur ce sujet,

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, lors de la passation de pouvoir entre l’ancien et le nouveau ministre de l’économie, M. Armand s’était estimé heureux « d’hériter d’un tel bilan Ce bilan, nous l’avons cet après midi devant nous, et les Français en subissent les conséquences ! L’étude de ce projet de loi de finances de fin de gestion laisse pantois. Comme nous l’avons déjà suffisamment souligné, le déficit s’est dramatiquement creusé, le dérapage atteignant près de 50 milliards d’euros en une seule année, et ce sans qu’aucune crise majeure ni aucun retournement soudain de l’économie soient venus justifier une telle dégradation. Lors de l’étude du projet de loi de finances pour 2024, nous avions alerté, à l’Assemblée nationale comme au Sénat, sur les prévisions optimistes et même, oserai je dire, irresponsables du Gouvernement. Le groupe Rassemblement national de l’Assemblée avait déposé une motion de censure contre le gouvernement d’alors, qui se refusait à présenter un projet de loi de finances rectificative.

Cette situation m’inspire un rappel historique. Il y a dix ans, le nouveau gouvernement grec découvrait les maquillages comptables laissés par son prédécesseur. Confronté à une situation critique, il lançait sans le vouloir son pays dans la plus grave crise financière et politique de son histoire, exposant aussi, ce faisant, les faiblesses congénitales de la zone euro.

comptes publics ont tenté de justifier cette contre performance en invoquant une prétendue élasticité nouvelle des recettes fiscales à la croissance. Ils ont affirmé qu’il était impossible d’anticiper, que tout avait été fait dans les règles, mais que des circonstances imprévues avaient empêché d’atteindre les objectifs fixés. Cette justification malhabile ne saurait tromper personne. Face à la dérive volontairement occultée des comptes publics, entreprises et ménages renoncent à investir. De plus, la situation économique apparaît en réalité bien plus dégradée que le Gouvernement ne le pensait. Les Français entendent déjà résonner l’écho des plans sociaux, de Michelin aux usines de foie gras du Périgord, en passant, dans le Nord, par ArcelorMittal. Le chômage refait lentement surface, et avec lui son lot de malheurs. Mes chers collègues, nous ne saurions donner quitus au Gouvernement : par ce projet de loi qui acte ses illusions et ses mensonges économiques, il ne propose que des économies éparses ou des reports importants qui grèveront le budget de l’année prochaine. Des recettes fiscales en chute libre, des dépenses imprévues, des reports compromettant l’avenir et une opacité coupable quant à la réalité budgétaire

ce texte nous fait entrer dans une sorte de faille spatiotemporelle : le passé et l’avenir se télescopent brutalement. Ce matin, nous nous projetions vers le futur en entamant la discussion générale du projet de loi de finances pour 2025, dont nous commencerons dans un instant à examiner les articles. Dans l’intervalle, nous repartons vers le passé, pour clore les comptes de l’exercice écoulé. Le projet de loi de finances de fin de gestion 2024 permet de dresser le constat d’un triple échec collectif : échec du redressement de nos comptes publics

trouve dans une situation déplorable. Cela s’explique d’abord et surtout par un demi siècle de légèreté budgétaire, au cours duquel le Parlement a cessé de croire qu’il est sain et même rationnel de voter un budget à l’équilibre. Pis, il s’est convaincu que notre économie se porterait mieux si nous nous endettions sans limites. Cette logique est aux finances publiques ce que la consommation débridée est à la préservation de la planète de même qu’un modèle de consommation infinie dans un monde aux ressources finies est un contresens, un modèle d’endettement infini dans un pays à la démographie déclinante et à la croissance morose est tout simplement une absurdité. OK, ! », diraient mes enfants. J’ai envie de dire plutôt : « KO, ! » Il faut changer de logiciel ; il faut changer de culture ; il faut changer de méthode. La génération qui exigera de ses responsables politiques qu’ils votent des budgets à l’équilibre est elle déjà née ? Je l’ignore, mais, en tout cas, je l’espère vivement. En attendant, si nous voulons redresser nos comptes, il est urgent de retrouver un horizon de projection souhaitable, en dehors du matraquage fiscal et de la dépense à gogo. l’échec de nos prévisions macroéconomiques. Le déficit public, cela a été rappelé, a dérapé de plus de 1 point de PIB depuis l’adoption du projet de loi de finances initiale. À qui la faute ? Le rapporteur général et le président de notre commission des finances ont conduit une mission d’information visant à identifier les failles dans la chaîne de responsabilité. Au delà de la mise en cause de telle ou telle personne, j’espère surtout que ces travaux seront l’occasion de formuler des propositions systémiques permettant d’éviter que de telles erreurs ne se reproduisent. À mon sens, c’est surtout l’inflation qui est en cause, elle qui nous fait perdre la raison et qui nourrit nos démons. Les prix augmentent ? Vite, dépensons plus pour protéger les particuliers et les entreprises, car, de toute façon, les recettes augmenteront à due concurrence et le déficit, rapporté à la richesse produite, n’explosera pas ! Encore raté… L’augmentation des recettes n’a pas suivi celle des dépenses et nous voilà renvoyés à notre incapacité à nous focaliser sur la réduction de notre déficit public

Pour tenter d’apporter une solution structurelle à ce triple échec, je vous ai proposé, mes chers collègues, de changer de méthode en renforçant la programmation pluriannuelle. Cette option n’a pas prospéré, je le déplore. Peut être n’était elle pas la bonne ? En tout cas, je reste convaincue qu’il n’est pas possible de continuer ainsi très longtemps. En attendant, le groupe Les Indépendants votera évidemment en faveur de ce budget de fin de gestion. ce texte ouvre des crédits pour éteindre le feu social et économique qui a pris en Nouvelle Calédonie et qui menace l’unité nationale. Ensuite, il ouvre des crédits pour payer les primes promises aux agents qui ont assuré la sécurisation des jeux Olympiques et Paralympiques. Lesdits agents ont contribué au rayonnement de la France dans le monde entier : nous le leur devons.

le testament. C’est le testament d’une gouvernance passée, qui n’a su ni anticiper ses ressources ni freiner ses dépenses. Et le coût des frais de succession est particulièrement élevé pour le gouvernement actuel, mais surtout pour la Nation et les Français une dégradation de 1,7 point du déficit public, soit un glissement de 50 milliards d’euros par rapport à la prévision initiale, et une impasse de 41 milliards d’euros sur les recettes publiques.

inférieure aux prévisions de l’ancien gouvernement, mais conforme aux estimations des principaux instituts, c’est grâce à l’investissement public et au commerce extérieur, et non, comme à l’accoutumée, grâce au moteur de la consommation en berne. On peut à ce titre regretter, et c’est un euphémisme, l’absence de collectif budgétaire au printemps. Elle marque une rupture démocratique que nul ne saurait accepter. Face aux prévisions de recettes erronées, visiblement insincères, auxquelles s’ajoute une insuffisance de freinage de la dépense malgré quelques expédients de régulation budgétaire, nous devons agir en responsabilité, à la fois, en faisant face à l’urgence, mais aussi en nous inscrivant dans l’anticipation pour préparer les nécessaires réformes structurelles. Soit Bercy a encore beaucoup plus de pouvoirs qu’on ne l’imagine, soit le politique a failli. Les deux hypothèses sont tout aussi inquiétantes l’une que l’autre. Quoi qu’il en soit, les gouvernements qui se sont succédé depuis 2022 ont mis en péril l’avenir de notre pays ; pis encore, ils ont peut être provoqué la crise démocratique que nous connaissons. La mission d’information sur la dégradation des finances publiques, conduite par notre commission des finances sous la houlette de son président, Claude Raynal, et du rapporteur général, Jean François Husson, a présenté ses conclusions accablantes voilà quelques jours. Après avoir remercié nos collègues pour leurs travaux, je veux m’y arrêter un instant, tant l’irresponsabilité budgétaire dont ont fait preuve les gouvernements en place d’octobre 2023 à septembre 2024 est grave, et tant le Parlement a été ignoré au cours de toute cette période. Il est désormais avéré que, dès décembre 2023, le gouvernement en place connaissait l’état critique des finances publiques. Il aurait donc dû réagir vigoureusement, et il ne l’a pas fait. Le fort risque de dégradation des recettes par rapport à la prévision était même identifié dès le 30 octobre 2023. Le double discours des ministres Bruno Le Maire et Thomas Cazenave est patent. Au premier semestre de 2024, le Gouvernement et le Président de la République ont donc refusé de présenter un projet de loi de finances rectificative, pourtant seul à même de redresser la situation, d’après le ministre des finances lui même. C’est une faute. Au total, rappelons le, le projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024 prévoit un écart en recettes par rapport aux prévisions du PLF pour 2024 de 41,5 milliards d’euros, dont 22,6 milliards d’euros proviennent d’un point de départ plus dégradé que prévu du fait des résultats de 2023. Le Gouvernement a pris des demi mesures, pas toujours assumées, et sans doute justifiées par des calculs politiques de courte vue. Avec le pari de la dissolution, pour lequel l’Histoire sera sans doute cruelle,

l’on pressent déjà dans ce PLFG. J’en viens donc à la promesse. C’est une promesse que nous n’avions pas connue depuis longtemps, la promesse d’un nouveau chemin, d’une sincérité budgétaire, d’un freinage de la dépense… Bien sûr, ce chemin sera long. La première marche proposée en 2025 est haute, mais nécessaire si nous voulons retrouver notre crédibilité sur la scène internationale et garantir notre souveraineté. Ce PLFG est un premier marchepied, avec un niveau de dépenses de l’État inférieur à ceux qui figurent dans la loi de finances initiale et dans la loi de programmation des finances publiques. Pour preuve, et je ne vais pas non plus les égrener, les diminutions de crédits portent sur la majorité des missions du budget général, tout en permettant l’accomplissement des missions jusqu’à la fin de l’année. Hors remboursements et dégrèvements, le montant des crédits annulés est supérieur de 1,9 milliard d’euros à celui des crédits ouverts. C’est la première fois depuis 2019 que le collectif budgétaire de fin d’année présente des économies par rapport à la loi de finances initiale. Dix missions connaissent des ouvertures nettes et vingt trois missions des annulations nettes en crédits de paiement.

Néanmoins, laissez moi m’étonner, pour ne pas dire plus, de l’incapacité de notre pays à honorer les loyers de nos gendarmeries auprès des bailleurs sociaux ou des communes. Heureusement, cela va être modifié – et cette mesure justifierait, à elle seule, le vote de ce PLFG. Mais, là aussi, quels errements dans la gestion ! Quelle insincérité ! La charge locative ancienne est une charge certaine. Un ménage, une entreprise, une collectivité qui ne l’intégrerait pas dans son budget serait sanctionné, rappelé à l’ordre. Mais l’État « d’un monde liquide » se l’était autorisé… Nous allons y remédier par notre vote, et je m’en réjouis. Face à un déficit budgétaire abyssal et historique à la fin de 2024, dont les gouvernements précédents portent seuls la responsabilité, un déficit subi par le Parlement et les Français, qui présente aujourd’hui un véritable risque de crise démocratique et institutionnelle, la nécessité de mesures de redressement conjuguant courage, responsabilité, rigueur, mais aussi espoir est bien certaine. monsieur le ministre, et nous voulons vous y aider, parce qu’il y va de l’intérêt général, de la place de la France et de l’avenir des Français. C’est la raison pour laquelle notre groupe adoptera ce PLFG amendé.

de la situation budgétaire pour l’année 2024, qui touche à sa fin. Il nous impose également un exercice d’introspection. Certains indicateurs traduisent une dynamique économique maîtrisée. La croissance économique, bien que modérée, demeure positive, avec une progression de 1,1 % du PIB. Le taux des prélèvements obligatoires diminue : 42,8 % en 2024 contre 43,2 % en 2023. L’inflation a été contenue à 2,1 %, contre 4,9 % en 2023. Les dépenses publiques s’établiront à un niveau inférieur de 6 milliards d’euros aux prévisions de la loi de finances initiale. Toutefois, Toutefois, l’année 2024 marque également une dégradation préoccupante de notre déficit public. Initialement estimé à 4,4 % du PIB, celui ci devrait finalement atteindre un Cette évolution n’est pas le résultat d’une dérive des dépenses, mais s’explique principalement par des recettes fiscales inférieures de 24,3 milliards d’euros par rapport aux prévisions. Un rapport de l’inspection générale des finances (IGF), publié en juillet 2024, éclaire ces difficultés. Il souligne que l’année 2023 a été marquée par des dynamiques atypiques l’élasticité des prélèvements obligatoires au PIB, qui mesure la croissance des prélèvements en rapport avec celle du PIB, a atteint une valeur de 0,42, bien inférieure à sa moyenne de longue période, proche de 1. Cette faiblesse, la deuxième de cette importance relevée depuis 1991, reflète les effets conjugués d’une inflation élevée liée à la crise énergétique de 2022 et du net ralentissement de la croissance de la masse salariale en fin d’année. L’IGF souligne ainsi la difficulté à anticiper les évolutions atypiques. Dans ce contexte, le groupe RDPI soutient pleinement les travaux menés par le Parlement et le Gouvernement pour améliorer la fiabilité des prévisions économiques et budgétaires. Nous saluons en particulier la mise en place, sous l’égide des ministres Antoine Armand et Laurent Saint Martin, d’un comité scientifique indépendant destiné à renforcer le pilotage des prévisions économiques et à mieux informer le Parlement. Bien que nous ne partagions pas toutes les conclusions de la mission d’information sur la dégradation des finances publiques, nous adhérons pleinement à son appel en faveur d’une meilleure association du Parlement, dans un esprit de transparence et de concertation, aux décisions relatives à la gestion des finances publiques. Nous pensons que la création de ce comité contribuera à éclairer nos débats. Je tiens également à souligner que l’action des gouvernements successifs, cette année, illustre une volonté constante de responsabilité budgétaire. Face à des prévisions macroéconomiques de plus en plus pessimistes, le gouvernement en place a agi tout au long de l’année 2024 pour compenser la moindre dynamique des recettes fiscales et limiter son impact sur le déficit. Ces efforts se sont traduits, d’une part, par un décret d’annulation de 10 milliards d’euros de crédits inscrits dans la loi de finances initiale pour 2024 et, d’autre part, par un gel supplémentaire de 16,5 milliards d’euros, visant à préserver des marges de manœuvre pour le gouvernement à venir.

Parallèlement, des fermetures stratégiques de crédits seront opérées, dans un souci de redressement des finances publiques. En somme, ce PLFG traduit la stratégie que nous devons poursuivre dans les années à venir : réduire le niveau de nos dépenses publiques de manière ciblée et concertée, afin de dégager des marges de manœuvre indispensables pour relever les défis du changement climatique, des aléas économiques et des enjeux de sécurité. Il nous invite également à rechercher des compromis et à œuvrer collectivement pour l’avenir de notre pays. C’est pourquoi, mes chers collègues, nous voterons ce texte de responsabilité et de vérité.

notre dette vient de s’alourdir de plus de 50 000 euros. Si encore ce creusement de la dette avait servi à l’investissement public et aux investissements d’avenir… Mais non ! Cet argent, malheureusement, est pour une grande part dilapidé dans le fonctionnement de l’État. Derrière ces chiffres vertigineux se cache une réalité préoccupante : nos méthodes de prévision budgétaire sont défaillantes. Comment expliquer un manque de 20 milliards d’euros de recettes qui n’avait pas été anticipé ? Monsieur le ministre, nous disposons d’une richesse inexploitée : les déclarations détaillées de nos entreprises sont une mine d’informations précieuses, que nous délaissons au profit de données macroéconomiques approximatives. Cette situation d’incertitude n’est plus tenable pour la deuxième économie de la zone euro. Face à des défis budgétaires majeurs, nous devons nous tourner vers l’intelligence collective de nos territoires et y prendre directement la température. rien ne peut justifier l’inaction face aux défis immédiats qui nous attendent. C’est là tout le paradoxe de notre situation : rejeter ce projet de loi de finances de fin de gestion pourrait apparaître comme irresponsable, mais l’adopter avaliserait des méthodes que nous nous refusons à cautionner. C’est là le dilemme ! Il nous faut regarder au delà des chiffres

aux valeurs démocratiques. C’est le premier acte de résistance que nous devons opposer aux ennemis de l’Europe. Très bien ! Je pense ensuite au soutien indispensable à la Nouvelle Calédonie. Nous ne pouvons laisser ce territoire dans la situation dramatique qui est la sienne aujourd’hui. Ne ternissons pas non plus la réussite des jeux Olympiques et Paralympiques, qui ont ébloui le monde par leur magie. Notre pays a démontré sa capacité à organiser un événement exceptionnel ; il doit maintenant mobiliser les moyens nécessaires pour boucler sereinement ce chapitre historique. citerai l’hébergement d’urgence pour nos concitoyens les plus fragiles, alors que l’hiver approche et que la précarité ne cesse de progresser. Ces engagements ne sont pas de simples lignes budgétaires. Ils incarnent notre pacte social, notre solidarité nationale et internationale. Derrière chaque euro de crédit se cache une réalité humaine. Reporter ces décisions au nom de la rigueur budgétaire serait non seulement une erreur politique, mais sûrement une faute morale. Car, si nous devons être intransigeants sur la gestion de nos finances publiques, nous ne pouvons l’être au détriment de nos valeurs fondamentales et de nos engagements les plus essentiels. C’est pourquoi, malgré nos inquiétudes légitimes sur notre endettement, malgré l’incurie de la gestion passée de nos finances publiques – vous n’y êtes pour rien, monsieur le ministre –, nous ne voulons pas nous opposer frontalement à l’adoption de ce texte. Mais cela ne signifie pas que nous cautionnons la gestion de vos prédécesseurs et les méthodes employées pour cacher l’ampleur réelle du déficit. Nous ne pouvons plus nous permettre cette navigation à vue, qui érode la confiance de nos concitoyens dans nos institutions. La confiance se mérite ; elle se construit sur la transparence de nos comptes publics et la fiabilité de nos prévisions. Il est temps de donner des gages concrets aux parlementaires et aux Français. Notre démocratie et notre cohésion sociale en dépendent.

urgent, je le dis, de fiabiliser nos prévisions de recettes et j’espère, monsieur le ministre, que conformément à vos engagements et à celui du ministre de l’économie, nous recevrons prochainement une documentation

d’euros. Jamais, face à une situation aussi critique, les responsabilités de ce dérapage n’ont été aussi peu assumées par les gouvernements qui en sont à l’origine, comme vient de le montrer la mission d’information

pluriannuels. À ces dérapages budgétaires s’ajoute un problème politique, puisque les mouvements de régulation budgétaire sont intervenus par voie réglementaire.

plus pressé. Il apparaît d’abord comme une nécessité, en raison des crédits qu’il permet d’ouvrir. Ces 4,2 milliards d’euros de crédits supplémentaires permettront de financer des mesures de soutien aux entreprises, aux forces de l’ordre, d’assurer le financement de nos armées ou encore de payer les suppléments de salaire de la fonction publique, notamment les primes liées aux jeux Olympiques et Paralympiques. Je profite de ce dernier point pour saluer la formidable réussite de cet événement historique, grâce à la mobilisation des moyens de l’État. Mais, et c’est là l’essentiel du présent PLFG, des efforts budgétaires importants sont réalisés. Les ouvertures de crédits sont en effet plus que compensées par l’annulation de 5,6 milliards d’euros de dépenses de l’État. En accord avec les ministères concernés, le Gouvernement a dégagé des économies sur l’aide publique au développement, la recherche et l’enseignement supérieur ou encore les engagements financiers de l’État. Ces annulations de crédits s’additionnent aux 5,8 milliards d’euros de moindres dépenses du budget général, permises par les 10 milliards d’euros de crédits annulés par le précédent gouvernement en février, une mesure de bon sens que nous saluons. projet de loi de finances de fin de gestion qui nous est présenté permet 7,4 milliards d’euros de moindres dépenses du budget général par rapport à ce qui était prévu en loi de finances initiale. C’est un fait particulièrement notable,

texte permet ainsi de stabiliser la dégradation des finances publiques, évitant que notre déficit ne s’envole à 6,2 % du PIB en 2024. Au vu de la situation budgétaire qui s’impose à lui, le gouvernement de Michel Barnier a donc fait le choix, dans l’urgence, de prendre ses responsabilités. C’est la première pierre sur le chemin du redressement des comptes publics, que concrétisera

et la viabilité budgétaire de notre pays, le groupe Les Républicains votera ce projet de loi de finances de fin de gestion, étape nécessaire au redressement des finances de la France. La discussion

qui va priver le plan Vélo de 250 millions d’euros pour l’année en cours, est un mauvais arbitrage budgétaire. Nous avons besoin de décarboner le secteur des mobilités, responsable de 29 % des émissions de gaz à effet de serre de notre pays. Ce n’est donc pas sur le développement des modes actifs de déplacement qu’il faut taper ; c’est sur ce qui va nous empêcher d’atteindre nos objectifs inscrits dans la stratégie nationale bas carbone, notamment pour Nous rejetons d’autant plus ces coupes qu’elles auront, une fois encore, un impact direct sur les collectivités. Rappelons que 400 projets d’aménagements cyclables sécurisés avaient été déposés par plus de 300 collectivités territoriales à la suite d’appels à projets gouvernementaux.

Les effets des dérèglements climatiques touchent notre pays de manière de plus en plus visible et concrète pour toutes et tous. Il y a urgence à changer de braquet. Nous proposons la suppression des alinéas 3 à 6 afin de garder un semblant de cohérence avec notre stratégie globale face à l’urgence climatique. Ne prenons pas aujourd’hui des mesures que nous regretterons demain

M. Simon Uzenat. Cet amendement vise à compenser l’extension de la prime Ségur aux organismes de formation en travail social. le 25 juin dernier, un accord a été agréé par le Gouvernement afin d’étendre cette prime à l’ensemble des professionnels non concernés dans le secteur sanitaire, social et médico social privé à but non lucratif, dont les organismes de formation en travail social.

sommes tous d’accord –, elle ne peut être imposée sans une discussion préalable avec les collectivités, dont la situation budgétaire est particulièrement fragilisée. Nous aurons l’occasion d’y revenir dans le cadre de

Les régions sont trop souvent laissées pour compte. Je ne reviendrai pas sur ce que l’État n’a pas fait pour elles ces dernières années, notamment au moment de la crise inflationniste. Nous maintenons donc cet amendement. Nous espérons que les membres de la majorité sénatoriale entendront raison sur ce sujet important

eux. Nous ne pouvons évidemment nous y résoudre. Je sais bien que je m’éloigne de l’objet de l’amendement, monsieur le ministre, mais je lance cet appel, en espérant que vous saurez y répondre, parce que nous avons plus que jamais besoin de ces structures pour accompagner les femmes qui subissent je vous remercie

En effet, comme cela a été rappelé, l’extension du « Ségur 2 » a eu lieu en milieu d’année 2024, avec effet rétroactif au 1 janvier, alors que tous les budgets des départements étaient votés. Christine Lavarde a évoqué, ce matin, la nécessité de respecter les règles quand on joue

je vous propose, par cet amendement de crédits, de compenser cette différence, de telle sorte que les départements ne se trouvent pas déséquilibrés dans leur exercice budgétaire. Quel est l’avis de la commission

les décisions de ce type, malheureusement habituelles de la part de l’État irresponsable, qui consistent à décréter des dépenses pour, dans le meilleur des cas, les financer avec de la dette pour ses opérateurs et, dans le pire des cas, comme ici, à ne pas les financer du tout, ce qui est absolument insupportable pour les collectivités. Cela dit, j’ai entendu

explication de vote. Je soutiens naturellement ces amendements, en cohérence avec celui que j’avais déposé et qui a malheureusement été rejeté par notre assemblée. Je dois vous avouer que ce n’est pas la première fois, depuis mon arrivée au Sénat l’année dernière, que je m’étonne de la façon dont les régions sont traitées. Pour moi, les choses sont relativement simples : le Sénat est la chambre qui représente les collectivités territoriales – toutes les collectivités territoriales

Et je pense qu’il est de bonne gestion de dire que les principes que nous édictons pour les départements doivent aussi s’appliquer pleinement aux régions, que nous parlions de libre administration ou d’autonomie fiscale et financière. Les régions ne vivent pas dans un monde parallèle

foulée du débat sur le Ségur, je vais évoquer la compensation aux départements de l’impact budgétaire, sur 2024, de l’augmentation de 4,6 % du RSA, qui est intervenue le 1 avril dernier.

exemples ! Si la revalorisation du dispositif RSA, notamment eu égard au niveau de l’inflation, est légitime dans un contexte social complexe, elle vient néanmoins se greffer à la longue liste de dépenses auxquelles les départements doivent désormais faire face

du fait de la baisse des DMTO, et à une progression constante de leurs dépenses de solidarité. De plus, cette évolution du RSA apparaît pérenne et structurelle. Elle devra, dès 2025, être absorbée par les départements sans pour autant être compensée par l’État, malgré l’engagement pris par ce dernier par le passé. Sur les 10,2 milliards d’euros de dépenses d’allocation du RSA, les départements auront un reste à charge de plus de 5 milliards.

certains pays – la Grèce n’est pas le seul exemple – n’ont pas été souverains dans le choix de leur budget, justement du fait d’un dérapage excessif de leurs finances publiques. Je crois que personne ici ne souhaite que ce soit le cas du nôtre. Nous avons donc un rendez vous

l’ensemble de la première partie du projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024. Je rappelle que, en application de l’article 42 de la loi organique du 1 août 2001 relative aux lois de finances, lorsque le Sénat n’adopte pas la première partie d’un projet de loi de finances de fin de gestion, l’ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté.

Ralentir la transition écologique dans les territoires aura des effets dramatiques sur le long terme, qui nous coûteront bien plus cher que les 500 millions d’euros économisés ici. La multiplication des catastrophes naturelles en France ne cesse de démontrer l’urgence d’agir, ainsi que la capacité des collectivités à mettre en

toutes et tous, du congrès des maires, qui s’est tenu la semaine dernière. Les maires ont clairement exprimé leurs inquiétudes quant à ces suppressions de crédits. Pour un certain nombre de dossiers, ils misaient sur ce levier de financement, dont ils ne pourront bénéficier

3 euros gagnés en cas de catastrophe naturelle. C’est pourquoi toute économie réalisée aujourd’hui sur le fonds Barnier se paiera trois fois plus cher dans les années à venir. Ce constat est d’autant plus vrai au regard de l’accélération du changement climatique et de la hausse

du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles de Mme Lavarde. Alors que 18,5 millions de Français sont concernés par les risques d’inondation et que 10,4 millions de maisons individuelles sont exposées au phénomène de retrait gonflement des argiles (RGA), il est nécessaire d’agir pour la protection de nos concitoyens et de les accompagner dans une démarche de prévention et d’adaptation au risque. Nous proposons donc, par cet amendement, d’augmenter les crédits consacrés à la prévention de 100 millions d’euros. Dans le contexte des inondations qui ont laissé tant de personnes sinistrées ces deux dernières années, il y a urgence

Cet amendement de notre collègue Patrick Chaize vise à abonder de 15 millions d’euros l’action n° 04 « Développement des postes, des télécommunications et du numérique » afin de rétablir les crédits de la mission « Aménagement du territoire En effet, la loi impose à La Poste le maintien des 17 000 agences postales, assurant ainsi un service public de proximité dans les territoires isolés. En contrepartie, le Gouvernement s’est engagé à verser à La Poste une compensation financière de 174 millions d’euros.

78 % de ces établissements estiment que ces difficultés financières auront un effet sur la qualité de leur prise en charge des personnes handicapées. Il vous est proposé, par cet amendement, de permettre à l’État de financer à hauteur de 50 % la part employeur, soit 25 % de la dépense totale de cette complémentaire santé. Cela représente un montant de 23 millions d’euros.

Financement structurel des écosystèmes d’innovation ». L’amendement n° 1, présenté par la commission des finances, tend à minorer les annulations de crédit sur la mission « Relations avec les collectivités territoriales » à hauteur de 70 millions d’euros.

comme chaque année, il nous revient d’examiner l’évaluation du prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne présentée dans le projet de loi de finances. Il s’agit d’un exercice incertain, dans la mesure où le montant inscrit dans le projet de loi de finances est seulement prévisionnel. Les négociations entre le Conseil et le Parlement européen autour du budget européen pour 2025 ont touché à leur fin ces derniers jours. Le 16 novembre dernier, ces deux institutions se sont accordées sur un montant de 199 milliards d’euros en crédits d’engagement et de 155 milliards d’euros en crédits de paiement. Ces deux institutions ont désormais jusqu’à la fin du mois pour approuver formellement l’accord intervenu. Le Conseil devrait l’adopter aujourd’hui même. Comme il est d’usage, le Gouvernement devrait déposer prochainement un amendement visant à tenir compte du montant du budget européen sur la contribution française. Je regrette, pour la clarté de nos débats, que nous ne disposions pas d’une évaluation révisée du prélèvement sur recettes (PSR). Pourriez vous, monsieur le ministre, nous indiquer quand sera déposé cet amendement ? Et quel serait le montant révisé de l’évaluation du PSR ? Une forte progression de la contribution française est attendue, ci étant estimée par la direction du budget à 30,4 milliards d’euros en 2026 et à 32,4 milliards d’euros en 2027. Si cette progression est en partie cyclique, la consommation des crédits se faisant plus marquée à mesure que l’on progresse dans le cadre financier pluriannuel, elle reflète le fait incontournable que la contribution annuelle moyenne de la France a fortement progressé, passant de 20,1 milliards d’euros par an entre 2014 et 2020 à 26,2 milliards d’euros par an entre 2021 et 2027.

Monsieur le ministre, un tel niveau de contribution est il soutenable dans le contexte budgétaire que nous connaissons ? Les négociations sur le prochain cadre financier pluriannuel commenceront l’an prochain ; quelle sera la position de la France ?

2020. Une telle mesure est indispensable pour notre pays. En effet, l’engagement financier de la France au titre de Next Generation EU est de l’ordre de 75 milliards d’euros. un défaut d’adoption de ces nouvelles ressources signifierait un surcroît de 2,5 milliards d’euros annuels sur la contribution française au budget de l’Union européenne à partir de 2028, qui s’ajouterait aux perspectives budgétaires préoccupantes que je viens d’évoquer. Monsieur le ministre, dans un contexte politique incertain, où la coalition qui gouverne l’Allemagne traverse une crise politique, quelles sont les perspectives d’adoption de ces nouvelles ressources propres ? Enfin, les sommes que j’ai évoquées ne visent qu’à financer les politiques publiques existantes de l’Union européenne. Or l’ancien président de la Banque centrale européenne (BCE), Mario Draghi, a fait état dans un rapport qui a fait grand bruit d’un déficit criant de compétitivité de l’économie européenne, nous appelant notamment à combler le fossé de l’innovation. L’actualité nous rappelle constamment que la compétition avec les puissances chinoise et américaine se fait chaque jour plus pressante. Draghi estime l’investissement nécessaire à un minimum de 800 milliards d’euros par an. Si le gros de ces investissements doit être endossé par le secteur privé, le rapport préconise, au vu des enjeux,

Cette bonne performance est une chance pour notre pays, ce plan finançant des projets très concrets, comme le chantier de la ligne C du métro toulousain ou la construction d’un nouveau bâtiment scientifique de l’Institut

Monsieur le ministre, cette bonne nouvelle ne doit cependant pas éclipser deux sujets d’inquiétude. Tout d’abord, si nous consommons les crédits du plan de relance européen, tel n’est pas le cas pour les crédits en gestion directe du budget de l’Union européenne, c’est à dire ceux qui sont directement exécutés par la Commission européenne, sans intervention des États membres. C’est particulièrement vrai pour la rubrique 1 du budget de l’Union européenne, consacrée à la recherche, à l’innovation et au numérique. Le taux de retour français sur cette rubrique est passé de près de 20 % en 2021 à environ 15 % en 2023.

Dans un contexte de finances nationales dégradées, alors que l’argent public se fait rare, nous ne pouvons pas nous permettre de nous priver de crédits européens. Le SGAE m’a indiqué que la France pouvait espérer bénéficier de 2 milliards d’euros de crédits européens supplémentaires. Il est donc impératif d’optimiser nos retours sur le budget de l’Union Enfin, j’appelle votre attention sur l’évolution de la contribution de la France. En 2028, doit commencer le remboursement du principal emprunt levé pour financer le plan de relance européen, dont le montant est de 750 milliards d’euros. En 2020, les États s’étaient accordés pour introduire de nouvelles ressources propres d’ici à 2026, afin de financer ce remboursement et d’éviter qu’il ne se traduise par un surcroît des contributions nationales.

Comme nombre d’entre vous, mes chers collègues, je rencontre très fréquemment des maires ou des présidents d’exécutifs qui me font part de leur désarroi quant à l’utilisation des fonds européens. Deux difficultés majeures sont fréquemment déplorées : la complexité de la procédure et le délai du versement. Les dernières données statistiques portant sur le sujet

manque encore de lisibilité. Les collectivités territoriales disposeront dans les années à venir de moins en moins de ressources, ou, à tout le moins, de plus en plus de besoins financiers. Leur faciliter l’accès aux fonds européens serait un réel coup de pouce

monsieur le ministre, mes chers collègues, le prélèvement sur recettes de la France au profit de l’Union européenne s’élève cette année à 23,3 milliards d’euros, soit une hausse de 7,9 % par rapport à 2024. cette tendance haussière n’est qu’un début. Dans un rapport publié le 25 juillet 2023, la Cour des comptes estime que la non adoption de ressources propres d’ici à 2028 contraindra la France

Cependant, le débat sur la définition de ces nouvelles ressources pour l’Union européenne s’enlise. Les nouvelles recettes envisagées seraient issues du système communautaire des quotas carbone, de revenus du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) et des bénéfices de certaines multinationales. Ces ressources sont injustes et volatiles et elles font la part belle au capital. Pourquoi ne pas s’accorder sur la taxation des transactions financières que propose la Commission européenne ? Cette ressource fondée sur la spéculation pourrait soulager la contribution des États membres. Il s’agit, mes chers collègues, d’une question prioritaire pour éviter que notre prélèvement n’explose ces prochaines années. grève nos marges de manœuvre, alors que la France est visée par une procédure de déficit excessif, car elle ne respecte pas les critères imposés par le carcan du pacte de stabilité et de croissance (PSC). La réponse du Premier ministre consiste en une cure d’austérité qui mettra à contribution les Français et leurs services publics.

Par ailleurs, la contribution de la France est aussi majorée par les rabais accordés à d’autres pays de l’Union européenne. Ce mécanisme antidémocratique est accordé par dérogation à certains États dont la contribution a été jugée excessive. L’Allemagne, l’Autriche, le Danemark, les Pays Bas et la Suède sont concernés. La France représente le premier contributeur à ces rabais : nous les finançons à hauteur de 1,5 milliard d’euros en 2025, soit 26,8 % du total. Nous pouvons donc légitimement douter de l’efficacité de notre contribution, d’un point de vue strictement comptable. La France est ainsi le deuxième pays contributeur net aux aux fonds européens, son solde net s’élevant à 9,3 milliards d’euros en 2023. Depuis 2017, la France a contribué à hauteur de 60 milliards d’euros en cumulé. Or elle n’est que le vingt deuxième bénéficiaire des dépenses de l’Union en 2023, avec 242 euros par habitant. que nous demeurons le premier pays bénéficiaire des fonds de la politique agricole commune. Mais en signant à tour de bras des accords de libre échange, la Commission européenne reprend d’une main ce qu’elle donne de l’autre. Nos agriculteurs en sont les premières victimes. le même temps, l’Union européenne durcit sa politique de lutte contre l’immigration et y met les moyens, au détriment de notre politique de réindustrialisation ou de transition écologique. Entre le cadre financier pluriannuel pour la période 2014 2020 et celui pour la période 2021 2027, les crédits alloués à la protection de l’environnement n’ont que légèrement augmenté, qui sont consacrés au contrôle des migrations et à la gestion des frontières ont explosé de plus de 700 %. De même, les crédits alloués aux investissements stratégiques européens ou pour l’interconnexion en Europe sont largement insuffisants : ils représentent 7 milliards d’euros, sur un budget total de 147 milliards La volonté de liquider Fret SNCF en est l’illustration. Nous devrions à l’inverse investir massivement pour faire advenir une nouvelle construction européenne axée sur un développement industriel en phase avec la préservation du vivant.

de répondre, une fois encore, aux critiques de ceux qui évaluent notre rapport à l’Europe en fonction de ce que cela nous rapporte, selon une logique comptable et transactionnelle fondée sur des sorties et des entrées,

bien moins que les avantages de la mutualisation des projets de recherche et d’innovation – on sait que seule l’Union européenne a la taille critique pour déployer des infrastructures et des programmes de niveaux comparables à ceux des États Unis ou de la Chine

pour nous de prendre la mesure des menaces et des exigences budgétaires qui se précisent pour l’Union et d’affirmer notre détermination commune à y répondre. Je pense à la menace de ne pouvoir faire face aux échéances de remboursement du plan post covid,

l’exigence, aussi, de financer les dépenses d’avenir. Le rapport Draghi montre combien nous devons axer notre politique sur trois axes prioritaires : la transition écologique, l’ambition industrielle et technologique

Comment faire aboutir ce cheminement décisionnel ? Comment gagner l’adhésion démocratique des peuples ? Je parle d’adhésion démocratique, alors que le scrutin européen a donné à l’extrême droite près d’un tiers de l’hémicycle

Ce n’est pas avec des nationalistes réactionnaires, pro Pouline, antisociaux, anti migrants délirants, sourds à la biodiversité et climatosceptiques que l’Union répondra aux menaces budgétaires grandissantes ni qu’elle traduira concrètement les orientations du rapport Draghi

était dû à des circonstances exceptionnelles, notamment des retards dans l’exécution des fonds de cohésion. En réalité, notre contribution au budget européen s’établit, depuis plusieurs années, autour de 25 milliards d’euros, contre environ 20 milliards d’euros dans les années 2010.

pluriannuel. Surtout, elles ont mis en lumière les limites du modèle financier de l’Union européenne. Car c’est bien là que réside le problème : un financement européen fondé quasi exclusivement sur les contributions nationales. D’un côté, nous demandons toujours plus à nos budgets nationaux, déjà sous tension. Pour la France, ce sont potentiellement 75 milliards d’euros supplémentaires à l’horizon 2058, soit 2,5 milliards d’euros de plus par an.

pour la PAC. En termes de retour par habitant, la France n’est que le vingt deuxième bénéficiaire des dépenses de l’Union européenne en 2023. Est ce satisfaisant ? Non, bien évidemment. Nous devons faire mieux, notamment sur des programmes comme Horizon Europe. Au delà des chiffres se pose une question plus fondamentale : l’Europe a t elle aujourd’hui les moyens de son ambition ? Nous le savons, les défis sont immenses : transition écologique, compétitivité industrielle, montée en puissance des tensions géopolitiques. Face à cela, continuer à fonctionner avec un budget limité et une dépendance quasi totale aux contributions nationales nous conduit à l’impasse. Aussi, que faire ? Tout d’abord, avancer réellement sur les ressources propres. Le rapport Draghi, publié en septembre dernier, est très clair pour sortir de cette dépendance, il faut un choc d’investissement, financé par des ressources autonomes. Les pistes existent : l’extension du marché carbone européen, le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières ou la taxation des multinationales sont autant de solutions concrètes, concrètes, déjà identifiées, mais leur adoption reste bloquée, souvent par une logique de « paquets » qui paralyse totalement les négociations. Il est temps de sortir de cette impasse. Ensuite, il faut envisager un nouvel emprunt européen commun. Nous y sommes favorables, à condition qu’il repose sur des ressources propres pérennes. Cet emprunt serait un outil puissant pour financer des investissements à long terme le renforcement de la défense et de la sécurité européenne, des infrastructures décarbonées pour accélérer la transition énergétique, des cofinancements pour les transports du quotidien, qui touchent directement nos concitoyens. Ce que nous défendons, c’est une Europe qui prend son destin en main, une Europe qui investit, non pas pour alourdir sa dette, mais pour créer des actifs durables et renforcer sa souveraineté. Il s’agit de bâtir une autonomie financière européenne, qui permette à l’Union européenne d’être à la hauteur de ses ambitions. Mes chers collègues, nous sommes à un moment charnière.

L’Europe, elle, reste empêtrée dans ses limites financières. Si nous ne réagissons pas rapidement, c’est non seulement notre position dans le monde qui est menacée, mais aussi notre capacité à garantir un avenir prospère à nos concitoyens. La révision du cadre financier pluriannuel intervenue en février 2024, qui a entraîné une augmentation de nos contributions, était une nécessité, mais, à terme, donner à l’Europe les moyens de ses ambitions ne pourra pas reposer uniquement sur nos budgets nationaux, qui ne peuvent tout porter seuls. Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain votera bien sûr cet article, mais il appelle également à un sursaut. Investir, se renforcer, redistribuer : tels sont les impératifs d’une Europe qui se veut écologique, souveraine, compétitive et protectrice. Ce sont les enjeux du futur cadre financier pluriannuel qui sera présenté par la Commission européenne en 2025. Nous ne pouvons pas nous contenter du. C’est à nous, parlementaires, de porter cette vision, pour que l’Europe redevienne ce qu’elle a toujours aspiré à être

Cette augmentation s’explique par la reprise du paiement des fonds de cohésion et par la faible hausse des ressources propres traditionnelles. Cette participation devrait d’ailleurs augmenter plus fortement encore dans les années à venir,

est confrontée à de tels enjeux mondiaux en matière de défense, de transitions, de recherche, d’innovation, de technologies telles que le quantique, le ou l’intelligence artificielle qu’il est impératif de lui octroyer les moyens d’y faire

de nombreux chantiers se profilent : la rationalisation des instruments existants, une plus grande flexibilité, sans compter la révision du prochain cadre financier pluriannuel ou la nécessité de se mettre d’accord pour trouver de nouvelles ressources propres. autant de sujets qui peuvent inquiéter quant au montant des futures contributions de la France. Toutefois, au delà de la reconstruction de nos industries, de notre engagement pour une économie plus durable, de la restauration de notre indépendance, il faut que l’Union européenne se pense et se considère comme puissance. Les conflits en cours à nos portes nous y obligent, et le résultat des élections américaines ne fait que confirmer la nécessité d’accepter notre rôle.

Nous devons donner l’impulsion à l’Union européenne dans le sens prôné par MM. Draghi et Letta. Démocratie, marché commun, climat, défense, autonomie stratégique : donnons nous les moyens d’être cette Europe forte. Nos peuples le méritent. Je crois, avec Julia Kristeva, que, « sans l’Europe, ce sera le chaos

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, avec un transfert de plus de 23 milliards d’euros, auxquels il faudra ajouter au moins 2 milliards d’euros net au titre des ressources propres traditionnelles, l’apport de la France au financement de l’Union européenne approchera les 26 milliards d’euros l’année prochaine.

les mieux dotées, au coude à coude avec la mission « Sécurités ». Bien sûr, si l’on prend en compte les retours des politiques européennes sur le territoire national, le solde repasse sous la barre des 10 milliards d’euros. N’oublions pas non plus que notre économie tire des bénéfices très substantiels de son intégration au marché unique : au minimum 120 milliards d’euros par an, soit 4 % de notre PIB, Il n’en reste pas moins que, à l’heure où l’état de nos finances nous contraint à un exercice budgétaire inédit, autoriser ce transfert de ressources va bien au delà du simple fait de satisfaire à une obligation contractuelle de la France. Il s’agit d’un geste financier fort, auquel le groupe Les Républicains souscrira en votant l’article 40 de ce projet de loi de finances. Il s’agit, surtout, d’un engagement politique sans équivoque vis à vis d’une Union européenne qui, au regard des grands bouleversements mondiaux, n’a jamais paru aussi nécessaire. face à la menace russe, qui perdure, face à la concurrence chinoise, qui s’intensifie, et face à la distance américaine, qui s’accroît, l’Europe est la bonne échelle, la seule en réalité qui nous donne une chance de rester à la table du monde, la seule qui nous permette de relever les défis de notre temps, qu’il s’agisse de l’enjeu énergétique et climatique, de la compétition technologique et stratégique ou encore de la gestion des flux migratoires. Pour remplir ces missions, l’Europe devra néanmoins apprendre à voir le monde tel qu’il se dessine, avec sa fragmentation croissante et ses rapports de force exacerbés. Elle devra aussi accepter de livrer de nombreuses batailles. La première d’entre elles sera économique, tant il est vrai que, sans prospérité, et donc sans moyens, aucun défi ne peut être relevé. être relevé. Or Enrico Letta et Mario Draghi l’ont rappelé : malgré sa force collective, l’Europe n’est pas aujourd’hui sur une trajectoire qui lui permettra d’être au rendez vous du XXI siècle. Leur constat est clair : l’Union européenne doit accélérer sa transformation économique. En premier lieu, ses politiques fondamentales devront se mettre au diapason de la nouvelle donne internationale. Certes, les principes d’ouverture commerciale et de libre concurrence devront rester au cœur du fonctionnement de notre marché. Cependant, face aux politiques industrielles agressives conduites à Pékin, à Washington ou ailleurs, leur mise en œuvre ne pourra rester en l’état : elle devra nécessairement évoluer pour intégrer de nouveaux concepts clés, par exemple celui de la réciprocité. Le traité Union européenne Mercosur en est un exemple douloureux. Puissance normative par excellence, l’Europe devra par ailleurs se rendre compte que, de l’agriculture aux technologies de rupture, la performance des entreprises passe aussi par l’efficacité réglementaire et par la retenue bureaucratique. Qu’elle passe, en outre, par des prix de l’énergie maîtrisés, donc par un marché de l’électricité révisé et une filière nucléaire confortée. Des réformes fondamentales devront donc être mises en œuvre. Elles seront toutefois insuffisantes si l’Europe n’investit pas massivement pour atteindre ses objectifs stratégiques en matière de défense, d’énergie, d’alimentation ou de maîtrise des frontières. Elles seront vaines si les capitaux nécessaires ne sont pas mobilisés pour stimuler l’innovation dans les technologies de demain : celles du spatial, du numérique ou de la transition écologique. Or, nous le savons tous, les financements nécessaires pour rester dans cette course sont colossaux. Alors que le prochain cadre financier pluriannuel devrait être mis en discussion l’année prochaine, ces besoins financiers relancent légitimement le débat sur la taille du budget européen. Mais ils relancent surtout l’idée de nouveaux emprunts Soyons toutefois réalistes : comment pourrait on envisager d’accroître nos dettes communes alors que, à ce jour, à peine un tiers des fonds du plan de relance post covid ont été consommés ? Comment accepter de s’engager sur de nouvelles émissions alors que, quatre ans après son élaboration, le plan de financement de Next Generation EU n’est toujours pas bouclé ? En effet, comme l’on pouvait malheureusement s’y attendre, la question des nouvelles ressources propres est encore en suspens. Je me rappelle que, déjà en 2009, à l’occasion de mon premier mandat de député européen, on évoquait l’urgence de mettre en place ces ressources propres… Certes, la Commission a fait des propositions en 2021, puis de nouveau en 2023. Mais, depuis lors, il s’est en réalité passé bien peu de choses au Conseil, et les divergences entre États membres restent particulièrement marquées. L’enjeu est pourtant fondamental : c’est d’abord une question de crédibilité pour l’Europe, mais c’est surtout une question financière, qui devient chaque jour plus urgente. En effet, si le remboursement des intérêts a déjà commencé, à des taux d’ailleurs bien plus élevés que cela avait été anticipé, le remboursement du principal, lui, commencera dans un peu plus de trois ans. À partir de là, ce seront au minimum 15 milliards d’euros supplémentaires qu’il faudra trouver chaque année. Si les nouvelles ressources propres devaient manquer à l’appel, cela se traduirait par un ressaut de la contribution française de plus de 2,5 milliards d’euros par an, soit une hausse d’environ 10 % du prélèvement sur recettes actuel. Dans de telles conditions, la charge que le budget européen ferait peser sur les finances nationales deviendrait une question encore plus sensible qu’elle ne l’est aujourd’hui. Il est donc essentiel de chercher les moyens d’en maîtriser la soutenabilité. Tout d’abord, bien sûr, il faut aboutir sur les nouvelles ressources propres. Puis, il faut mettre enfin sur pied une union des marchés de capitaux capable de mobiliser l’épargne inexploitée, donc de suppléer en partie aux fonds publics européens pour le financement des investissements d’avenir.

voilà une vingtaine d’années, près de 17 % des dépenses européennes étaient effectuées sur le territoire français ; aujourd’hui, ce taux de retour est tombé à 11,5 %. %. Certes, la composition de l’Union européenne a beaucoup changé depuis le début des années 2000, ce qui explique cette évolution défavorable. Il n’en reste pas moins qu’il y a là des gisements de ressources inexploités qui, en ces temps de disette budgétaire, doivent impérativement être mieux identifiés et mieux captés par notre pays. Cette recherche d’efficacité, en somme, devra plus que jamais devenir, dans les années qui viennent, le maître mot de la France, comme celui de l’Europe.

pour l’année 2025, la contribution française à l’Union européenne s’élèvera à 23,3 milliards d’euros, marquant une augmentation de 1,7 milliard d’euros par rapport à la loi de finances pour 2024.

Ce montant global comprend notamment les subventions allouées au titre de la politique agricole commune : 9,5 milliards d’euros pour notre secteur agricole, afin de favoriser notre souveraineté alimentaire, d’assurer un revenu à nos agriculteurs et de répondre au mieux aux enjeux du changement climatique. La contribution nette de la France à l’Union européenne pour 2025 sera de plus de 7 milliards d’euros. À cela s’ajoutent À cela s’ajoutent environ 2 milliards d’euros issus des ressources propres traditionnelles, principalement des droits de douane prélevés sur les importations de pays tiers, nets des frais de perception, portant ainsi la contribution nette totale à 9 milliards d’euros. Des hausses significatives du prélèvement sur recettes sont prévues pour les années 2026 et 2027 ci sera porté à 30,4 milliards d’euros puis à 32,4 milliards d’euros. C’est pourquoi, monsieur le ministre, il est impératif d’œuvrer à l’adoption de nouvelles ressources propres pour l’Union européenne, afin de limiter ces augmentations futures. En effet, l’engagement financier de la France au titre de l’emprunt Next Generation EU avoisine 75 milliards d’euros, et cet emprunt est censé être remboursé par le biais de nouvelles ressources propres. À cet égard, la Commission européenne a proposé en 2023 plusieurs a proposé en 2023 plusieurs mécanismes pour garantir un financement durable. Une part accrue des recettes du système européen d’échange de quotas d’émission de CO2 constituerait un premier volet de financement, dont 30 % seraient affectés au budget de l’Union européenne dès 2028. Le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, qui vise à prévenir les fuites de carbone et à égaliser les coûts pour les importations extraeuropéennes, pourrait également rapporter 1,5 milliard d’euros annuels à l’Union La taxation des bénéfices résiduels des multinationales dans le cadre de l’accord OCDE G20 sur la fiscalité internationale représenterait une contribution supplémentaire d’euros et 4 milliards d’euros par an. Enfin, la Commission propose une ressource temporaire fondée sur l’excédent brut d’exploitation des entreprises nationales, qui rapporterait annuellement 16 milliards d’euros entre 2028 et 2030 pour répondre à des besoins ponctuels. Il est absolument nécessaire de parvenir à un accord sur la question des nouvelles ressources propres. Le groupe RDPI y sera attentif. Nous voterons évidemment cet article

Pour 2025, cette contribution suit la trajectoire de hausse, après deux exercices budgétaires européens qui s’étaient soldés par une sous exécution des dépenses, trajectoire tracée par le cadre financier pluriannuel 2021 2027, lequel a été entériné par la loi du 18 décembre 2023 Notre participation par le prélèvement sur recettes s’établit cette année à 23,3 milliards d’euros. Globalement, l’ambition exprimée par l’Union européenne au travers de son budget porte la marque des enjeux actuels du continent. la relance économique qui a suivi la crise de la covid 19 a conduit les membres à s’accorder sur le plan Next Generation EU à hauteur de 750 milliards d’euros. Sur ce point, d’ailleurs, il demeure des questions relatives à son remboursement je nous invite à la vigilance pour éviter que cela ne pèse sur les contributions des États membres. Cherchons plutôt vers de nouvelles ressources propres qui s’ajouteraient aux ressources La création d’une taxe carbone aux frontières ou la mise en place d’une contribution des géants du numérique sont des mesures soutenues depuis longtemps par le RDSE. Dans cet effort commun, il faut également mentionner le soutien à la défense de l’Ukraine face à l’agression de la Russie, guerre qui conduit l’Europe à financer fortement son indépendance énergétique vis à vis du gaz russe. Ces dépenses constituent des investissements dans la coopération européenne. L’adoption par le Sénat de cet article 40, que l’Assemblée nationale a rejeté dans les circonstances que l’on sait, ne doit pas nous exonérer d’une réflexion large sur l’état de l’Union européenne et ses perspectives d’évolution. En effet, les défis auxquels nous faisons face appellent sans doute des réflexions structurelles face à la défiance, le renforcement du parlementarisme européen est indispensable pour légitimer de nouvelles dépenses qui doivent être menées au niveau communautaire. Le renforcement de notre souveraineté politique et budgétaire est pressant au regard de l’agenda politique outre Atlantique. Je pense notamment à l’insuffisance des crédits alloués à la défense européenne à l’heure où la prochaine installation du président élu américain nous contraint cette question : devons nous avoir la capacité de nous défendre sans les États Unis ? Cette défense doit être fondée sur une souveraineté du continent en matière d’armement, au travers de commandes publiques européennes et d’investissements dans les lignes de production. Je pense également au défi climatique : les investissements pour atteindre les objectifs d’ici à 2050 sont estimés à 3 600 milliards d’euros par la Commission européenne. La mutualisation de ces crédits permettra leur soutenabilité.

Ainsi, cette participation de la France au budget de l’Union européenne doit recevoir toute notre attention et faire l’objet de toute notre vigilance, mais, en l’état, elle renforce notre capacité à faire face aux enjeux contemporains. Pour toutes ces raisons, le groupe RDSE votera dans

Cet ajustement financier permettrait également de recentrer les ressources nationales vers nos objectifs vitaux, comme la réduction de la dette publique et le soutien aux services publics. L’amendement

projet de loi de finances pour 2025 dénombre 474 dispositifs fiscaux dérogatoires classés comme dépenses fiscales. Le coût des dépenses fiscales pour 2025 est estimé à plus de 85 milliards d’euros.

En dernier point de l’ordre du jour du jeudi 12 décembre, il demande d’inscrire la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à prolonger la dérogation d’usage des titres restaurants pour tout produit alimentaire.

Acte est donné de ces demandes. Pour chacun de ces textes, nous pourrions fixer le délai limite pour l’inscription des orateurs des groupes la veille, à